J'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein des éventuelles commissions mixtes paritaires chargées d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi relatif à l'énergie et au climat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

Cette promotion et les nouvelles responsabilités qui l'accompagnent vous offrent désormais de nouvelles compétences pour passer des intentions aux actes. Vous avez récemment promis que la ligne de fret Perpignan-Rungis

! On conviendra qu'en plus d'être économiquement absurde, cette situation est écologiquement irresponsable. Votre champ de compétence vient de s'élargir considérablement, madame la ministre. Vous allez pouvoir mettre en oeuvre une solution un peu plus sérieuse pour maintenir cette ligne et cesser de faire circuler un train fantôme. Avec

la priorité du quinquennat. Je mesure l'ampleur des défis que nous aurons à relever et je ne doute pas que nous pourrons y travailler ensemble. Ma feuille de route est de poursuivre et d'accélérer les transformations en cours.

Je sais que votre commission l'a complété dans une logique constructive. Le Gouvernement sera amené à déposer quelques amendements, sur des sujets essentiellement techniques. Je forme le voeu que nous puissions poursuivre

Ce plan prévoit l'injection d'hydrogène dans les réseaux comme levier de flexibilité et de stockage, facilitant l'intégration des énergies renouvelables électriques intermittentes dans le mix énergétique. Le présent amendement vise donc à inscrire dans le code de l'énergie un objectif de développement du recours à l'hydrogène bas-carbone et renouvelable, pour les usages non seulement industriels,

Cet objectif reste d'ailleurs inférieur aux projections réalisées dans le cadre du plan de déploiement de l'hydrogène pour la transition énergétique, qui prévoit la production d'environ 450 000 tonnes d'hydrogène bas-carbone et renouvelable à l'horizon 2028. L'amendement n°

dans la consommation totale d'hydrogène à l'horizon 2030. En outre, cet amendement ne supprime pas l'objectif relatif à l'hydrogène industriel, qui garde toute sa pertinence. L'amendement n° 23, à favoriser l'utilisation de l'hydrogène dans les transports. Sa finalité est compréhensible, puisque le recours à l'hydrogène dans le domaine des mobilités constitue l'un des axes du plan de déploiement de l'hydrogène et figure parmi les objectifs du projet de PPE.

pour remédier aux tensions sur le système électrique. Le pilotage de la consommation de pointe par les effacements présente des atouts importants et multiples pour la transition énergétique : économies d'énergie, contribution à la sécurité d'approvisionnement. Or, malgré ces atouts majeurs, les effacements sont aujourd'hui très insuffisamment développés.

aussi bien au niveau de la production qu'à celui de la consommation. Je suis certes favorable au développement des effacements de consommation ; néanmoins, en se focalisant sur la seule demande,

Dans le cadre des objectifs de la politique nationale énergétique, il est essentiel d'apporter un soutien particulier au développement du fret ferroviaire et fluvial, afin de pouvoir réduire les émissions de gaz à effet de serre et atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050.

en 2017, le transport ferroviaire et fluvial de marchandises ne représentait que 11,5 % du total, bien loin de cet objectif initial de 25 % fixé par la loi.

actuellement en discussion, qui prévoit d'améliorer l'efficacité des transports de marchandises afin de renforcer la compétitivité des territoires et des ports, d'accélérer le report modal et de diminuer l'impact environnemental du fret. Nous proposons de compléter l'article L. 100-4 du code de l'énergie et de fixer dans la loi cet objectif ambitieux de soutien au fret ferroviaire et fluvial. Permettez-moi, madame la ministre, de vous dire

Par ailleurs, on notera que l'article 51 du projet de loi d'orientation des mobilités, en cours d'examen, prévoit déjà la définition d'une stratégie pour le développement du fret ferroviaire sera plus complète que moi sur ce point. Enfin, les aspects énergétiques du transport pourront être abordés dans le cadre du volet de la PPE portant sur la réduction de la consommation énergétique et des objectifs relatifs au carburant de la loi quinquennale.

notamment pour le transport de marchandises. Comme l'a dit M. le rapporteur, l'un des cinq programmes prioritaires de la programmation des infrastructures qui fait partie de la loi d'orientation des mobilités prévoit d'investir 2,3 milliards d'euros, dans les dix prochaines années,

que « ses performances en matière de sûreté nucléaire sont en retrait par rapport à l'appréciation générale que l'ASN porte sur EDF. Dans le domaine de la sûreté nucléaire, l'ASN constate que la qualité des opérations d'exploitation s'est détériorée par rapport aux années précédentes, ce qui se traduit par la déclaration de nombreux événements significatifs pour la sûreté, dont quatre classés au niveau 1 de l'échelle INES. » Il nous faut

telles modifications ne sont pas utiles au regard du droit existant. En effet, le code de l'énergie prévoit déjà l'obligation de fixer dans la PPE, pour la seconde période de cinq ans qu'elle couvre, des options hautes et basses en fonction des hypothèses envisagées. Le pouvoir réglementaire peut donc tout à fait moduler les objectifs inscrits dans la PPE pour prendre en compte la sûreté nucléaire. Au demeurant, c'est déjà ce qui se passe en pratique, puisque, dans le cadre du projet de PPE, le Gouvernement se réserve la possibilité de demander la fermeture de réacteurs supplémentaires à EDF sous conditions assez strictes, notamment pour faire face à une décision éventuelle de l'ASN

a prévu qu'une feuille de route des opérations de démantèlement des installations nucléaires lui soit annexée. La commission émet donc un avis défavorable sur ces amendements.

est à Mme la ministre. L'alinéa 32 vise à prévoir, en annexe à la programmation pluriannuelle de l'énergie, une feuille de route relative aux opérations de démantèlement des installations nucléaires. Si le succès du démantèlement de ces installations est essentiel, une telle feuille de route n'a pas vraiment sa place en annexe de la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui doit rester un document de politique énergétique. Les éléments relatifs aux installations nucléaires sont par ailleurs débattus dans le cadre du Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, qui fait actuellement l'objet d'un débat public. De plus, le choix des réacteurs à fermer est d'abord du ressort de l'exploitant des centrales nucléaires. Les désigner dans une annexe à la PPE serait de nature à prolonger les discussions sur ce document et à introduire des retards préjudiciables pour la politique énergétique.

la commission a refondu les feuilles de route annexées à la PPE en les ciblant sur l'essentiel : la rénovation thermique, qui découle d'une directive européenne du 30 mai 2018, le démantèlement des installations nucléaires, sur proposition de la rapporteure pour avis de la commission du développement durable, l'association des citoyens et des collectivités à la production d'énergie renouvelable, sur proposition de Mme Préville et de plusieurs de ses collègues. Il est d'ailleurs regrettable, madame la ministre, que le Gouvernement envisage de revenir sur ces deux derniers documents qui concourent à renforcer l'information du grand public sur des sujets essentiels. La commission émet un avis défavorable pour avis. La PPE a vocation à fixer, énergie par énergie, les grandes orientations de la politique énergétique française. Pour ce faire, elle précise aussi les moyens mis en oeuvre pour atteindre ces objectifs. comment pouvez-vous prévoir de ramener à 50 % la part du nucléaire dans le mix énergétique en 2035, donc engager la fermeture de quatorze réacteurs, sans préciser quels moyens vous allez mettre en oeuvre pour atteindre cet objectif ?

accepte de discuter de la réduction de la part du nucléaire de manière assumée, ce qui n'a pas toujours été le cas- je me suis un peu enflammé hier, vous n'étiez pas encore là, en parlant de moment « historique

Je rappelle qu'il prévoit l'ajout d'une annexe sur la stratégie pour le développement des projets de production d'énergie renouvelable dont tout ou partie du capital est détenu par les citoyens, les collectivités territoriales et leurs groupements.

plusieurs. L'amendement n° 174 vise à ajouter en annexe de chaque programmation pluriannuelle de l'énergie une feuille de route de réduction de la consommation énergétique du transport aérien

2050 et que la France est en pointe dans l'innovation technologique et industrielle dans le secteur aérien, il paraît nécessaire d'accompagner le verdissement de ce dernier.

très importante de polluants atmosphériques, notamment du soufre, de l'oxyde d'azote et des particules fines. La réglementation internationale en vigueur, bien qu'elle exige l'utilisation de carburants

Le carburant qui sera utilisé massivement à partir de 2021 contiendrait toujours 500 fois plus de soufre. Une feuille de route permettant de suivre l'évolution de la consommation énergétique dans ces deux secteurs serait tout à fait pertinente et intéressante.

Enfin, et surtout, ces transports n'étant pas clairement limités dans l'amendement aux sociétés ayant leur siège social en France ou assurant des liaisons à destination et au départ de notre pays, le dispositif pourrait conduire à évaluer la consommation énergétique de sociétés étrangères.

La PPE, comme vous le savez, comprend déjà un volet « transport », avec la stratégie de développement de la mobilité propre, qui inclut tous les modes de transport. Par ailleurs, les transports aérien et maritime les transports aérien et maritime domestiques sont bien inclus dans les émissions territoriales de la France, mais ce n'est pas le cas du transport international. Au regard de la croissance actuelle et attendue du secteur, le Gouvernement a été favorable à la définition du budget carbone additionnel pour les transports aérien et maritime internationaux, afin qu'ils soient bien inclus dans nos stratégies. Je souligne également que la loi d'orientation des mobilités prévoit la remise

complexifierait le contenu de la PPE. Par ailleurs, il est pour partie satisfait par les dispositions introduites à l'article 1 en commission. D'une part, la « valorisation de la biomasse à des fins énergétiques » et la « production simultanée de chaleur et d'électricité » ont été inscrites parmi les objectifs de la politique énergétique.

est à M. Roland Courteau. Cet amendement vise à faire passer la programmation pluriannuelle de l'énergie du niveau réglementaire à l'échelon législatif, en prévoyant une loi de programmation. Certes, il ne nous a pas échappé que l'article 1 A, introduit par les députés, prévoit désormais l'adoption tous les cinq ans d'une loi fixant les objectifs et les priorités d'action de la politique énergétique nationale. C'est une avancée, et nous nous félicitons que le Parlement puisse de cette manière être associé à la programmation pluriannuelle de l'énergie grâce à une loi quinquennale. Notre ambition est toutefois beaucoup plus large,

avec la loi quinquennale créée par l'article 1 A, qui permet au législateur de fixer, notamment, les priorités d'action dans le domaine de l'énergie. Au demeurant, il est moins ambitieux que cette loi, dont le champ s'étend également à la politique climatique. En outre, tel qu'il est rédigé, cet amendement conduit le législateur à se prononcer, non seulement sur les priorités d'action, mais aussi sur le contenu même de sept volets très techniques, qui relèvent clairement du domaine réglementaire. Enfin, il nie la spécificité de la Corse et des collectivités d'outre-mer, en tendant à supprimer l'existence des huit PPE distinctes et à retirer une compétence à certaines collectivités où la PPE est intégrée au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. Plutôt que de créer une nouvelle loi, il est préférable de tout mettre en oeuvre pour appliquer la loi quinquennale, d'autant que la commission l'a renforcée par huit amendements. C'est donc à une véritable inversion

notre production électrique. À titre de comparaison, les énergies renouvelables en totalisent moins de 20 %. Alors que les gouvernements successifs nous assurent que la transition énergétique est enclenchée et que nous allons, dans les années à venir, nous tourner davantage vers les énergies vertes, force est de constater que les efforts sont pour le moment timides. Il semble ainsi évident que l'ouverture de nouvelles centrales nucléaires tuerait dans l'oeuf toute ambition en matière d'énergie verte. Le présent amendement vise donc à introduire dans la loi l'interdiction de l'ouverture de nouvelles centrales nucléaires, afin de rendre effective la volonté affichée par l'exécutif de produire des énergies plus propres. Nous ne prenons pas à la légère les nombreux emplois que représente encore aujourd'hui le parc nucléaire français, tout comme nous ne nions pas que cette énergie est décarbonée. ne pouvons toutefois accepter le risque dû à l'exploitation de cette énergie pour nos concitoyens. Personne ne veut qu'un Tchernobyl ou un Fukushima se produise sur notre territoire. Si développé soit-il, le savoir-faire français ne peut assurer un risque zéro lorsqu'il s'agit de manipuler de la matière radioactive. Il est temps de passer à un modèle énergétique véritablement durable. Le présent amendement ne peut que nourrir cette dynamique. Quel

ce qui nuirait à la sûreté nucléaire ainsi qu'à la réalisation concrète de la trajectoire de réduction de la production nucléaire à 50 % de la production d'électricité d'ici à 2035, comme le prévoit l'article 1. De surcroît,

Par ailleurs, comme cela a été explicité dans le projet de PPE, le Gouvernement souhaite laisser ouverte l'option de construction de nouveaux réacteurs. Un rapport sur le sujet doit être remis mi-2021. L'avis du Gouvernement est donc défavorable, afin de laisser ouverte cette option et de permettre la mise en exploitation de la centrale

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues,

qui fixera les priorités d'action pour répondre à l'urgence climatique et écologique, en précisant, entre autres, les objectifs de développement des énergies renouvelables et de diversification du mix de production d'électricité. Comme vous le savez, l'Agence a mené des études en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion, afin d'évaluer la faisabilité de l'autonomie énergétique de ces territoires à l'horizon 2030. Elle y a donc étudié le potentiel d'énergies renouvelables disponibles et mobilisables, arrivant à la conclusion qu'un mix électrique composé de 100 % d'énergies renouvelables était techniquement possible. Selon ses estimations, la production annuelle d'électricité à partir d'énergies renouvelables variables représenterait entre 35 % et 53 % de la production totale en 2030 pour la Guadeloupe et La Réunion, quand elle serait comprise entre 58 % et 73 % en Martinique. Pour ce faire, il sera nécessaire de solliciter de manière très significative les potentiels en énergies renouvelables. Or les projets d'énergies marines renouvelables sont arrêtés ou en attente dans ces trois territoires, dont le projet NEMO en Martinique, suspendu depuis plus d'un an. pourtant permettre à la Martinique d'accroître substantiellement son indépendance énergétique en alimentant 35 000 foyers supplémentaires en énergie renouvelable. Le constat est le même s'agissant de La Réunion, avec le désistement de Climabyss, filiale d'Engie, en 2016, ou encore avec l'arrêt du projet d'énergie houlomotrice CETO en 2014. La situation est quant à elle un peu différente en Guadeloupe concernant le projet d'éolien offshore, puisque les études nécessaires au lancement de constructions n'ont toujours pas été engagées ! Pourtant, l'énergie thermique des mers, qui consiste à exploiter le différentiel de température des océans entre les eaux de surface et les eaux profondes afin de produire de l'électricité, est une alternative plausible et crédible aux énergies fossiles dans les outre-mer. Madame la ministre, je conclurai en rappelant que les intentions sont toujours bonnes, mais que les actes sont tellement meilleurs ! La parole Poadja, sur l'article. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je souhaite prendre rapidement la parole sur cet article, le seul qui mentionne les outre-mer, alors que c'est dans nos territoires que les enjeux de la transition énergétique et du climat sont les plus importants ! Les outre-mer abritent des réserves de biodiversité exceptionnelles, qui sont directement menacées par le changement climatique. Ce sont également des territoires particulièrement polluants et pollués, puisque l'essentiel de leur énergie provient des énergies fossiles : charbon, fioul, gasoil et gaz naturel. Ce sont enfin les plus exposés aux risques majeurs associés au dérèglement climatique : la multiplication des cyclones, la montée inquiétante du niveau des océans, l'augmentation des températures de l'air, mais aussi des océans, et leurs conséquences désastreuses sur la biodiversité ... Il me semble donc important de rappeler que, même s'ils pèsent peu sur les statistiques nationales, les outre-mer ne doivent pas être les oubliés de ce projet de loi. Au contraire, nous comptons sur vous pour leur donner une place centrale dans sa mise en oeuvre. La

pour faire de la transition énergétique un processus démocratique et partagé. En effet, cet article prévoit de transformer la PPE en une loi de programmation, sur le modèle, notamment, des lois de programmation des finances publiques. Il apparaissait inconcevable, voire surréaliste, Parlement ne soit pas saisi d'un tel document, compte tenu de ses enjeux environnementaux, financiers, sociaux ou en termes d'aménagement du territoire. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 part prévu la saisine de nombreuses instances, laissant cependant le Parlement quasi absent des discussions autour des orientations stratégiques de la France en matière d'énergie. Jean-François Husson et moi-même souhaitons que ces lois de programmation soient l'occasion de fixer des objectifs plus réalistes à moyen terme, afin que la transition énergétique ne soit pas seulement une addition de bons sentiments et d'injonctions pour les générations futures, mais qu'elle fixe également une liste d'objectifs pragmatiques et réalistes pour les générations d'aujourd'hui.

une loi tous les cinq ans pour fixer les objectifs d'action et la marche à suivre, afin de répondre à l'urgence climatique et écologique. À l'occasion de cette prise de parole,

les objectifs intermédiaires de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l'empreinte carbone de la France, les objectifs de réduction de la consommation d'énergie par secteur d'activité, les objectifs de développement des énergies renouvelables pour l'électricité, la chaleur et le gaz, ainsi que les objectifs de diversification du mix de production d'électricité. Le présent amendement vise à garantir que cette révision périodique s'inscrive pleinement dans la lignée des engagements que la France a pris dans le cadre de l'accord de Paris, des objectifs européens dans ce domaine et des trajectoires définies par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Il tend à clarifier ainsi l'objet de cette loi, dont le but est bien de fixer les priorités d'action

C'est pourquoi nous proposons d'intégrer les accords-cadres de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques dans la loi quinquennale, afin de nous inscrire dans le cycle de révision des engagements pris par la France dans le cadre de l'accord de Paris, et dans la lignée des objectifs européens. La parole

Sur le premier plan, il nous semble essentiel que l'accord de Paris constitue une boussole pour les futures lois de programmation énergétique, ce qui répond à une problématique très claire : faire en sorte que ces lois s'inscrivent dans les engagements internationaux de la France et ne visent qu'à fixer les moyens d'arriver à l'objectif fixé en décembre 2015. ne pourrions pas comprendre, alors que l'urgence climatique se fait de plus en plus pressante, que la France, au détour d'une loi purement nationale, revienne sur ses ambitions au prétexte que son contexte particulier l'exige. et c'est une des failles de l'accord de Paris, mais aussi, avant lui, du protocole de Kyoto, le caractère contraignant de ces accords est tout relatif. Certes, l'accord de Paris prévoit un certain nombre de mesures obligatoires, qui ouvrent la voie à des recours juridiques. Toutefois, en l'absence de mécanismes de contrôle et de sanctions, il paraît bien difficile de faire appliquer ce droit.

Inscrire dans la loi ces ambitions, c'est conforter la portée juridique des engagements français en matière de lutte contre le réchauffement climatique et pour une consommation énergétique responsable et raisonnable. Ce n'est pas en recevant les ONG de l'Affaire du siècle ou en pérorant « » que l'État s'engagera ! Le Président de la République a déclaré en mars dernier que la bataille climatique ne se jouerait pas sur le terrain judiciaire. Pourtant, c'est bien par ce biais que le Gouvernement pourrait être contraint à agir, comme un de ses prédécesseurs en 2009 dans l'affaire des algues vertes bretonnes, ou comme les Pays-Bas, sommés d'intensifier leur lutte contre le réchauffement climatique à la suite d'une saisine judiciaire de la fondation Urgenda. Si l'État n'est pas le seul responsable du changement climatique, il y participe par la pollution qu'il provoque et par les actes qu'il prend ou ne prend pas.

face au retard pris, préfère changer l'objectif plutôt que de le mettre en oeuvre avec les moyens nécessaires. La

sans qu'il faille les mentionner explicitement, puisque ceux-ci sont placés au-dessus d'elle dans la hiérarchie des normes. En effet, l'article 55 de la Constitution dispose que « les traités

est à Mme la ministre. Le présent amendement vise à consolider le nouveau dispositif d'élaboration de la politique énergétique et de la loi quinquennale. Il s'agit

les CEE, étant un moyen et non pas un objectif de notre politique énergétique et climatique. Il est également proposé d'adapter d'adapter la procédure de consultation sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE, en tenant compte du fait que, désormais, les grands objectifs seront définis dans une loi.

Cette modification constitue une avancée positive pour la filière, qui a besoin d'une visibilité à long terme pour se structurer et se développer. Les efforts de recrutement et de formation sont importants pour permettre la mise en place d'une filière à la hauteur des objectifs du dispositif, et qui puisse garantir la qualité des travaux réalisés. Par ailleurs, ces travaux nécessitent des matériaux et des équipements- équipements de chauffage, isolants, etc. dont la disponibilité doit faire l'objet d'une programmation à long terme. Il est proposé que la loi précise le niveau d'obligations pour deux périodes de cinq ans, afin de permettre à l'ensemble de la filière de bénéficier en permanence d'une visibilité suffisante. Le niveau de la seconde période serait réévalué dans le cadre de la loi quinquennale suivante.

un tel débat devait avoir lieu, il ne devrait pas se tenir concomitamment à l'examen du projet ou de la proposition de loi par le Parlement, mais il pourrait intervenir avant ou après le débat parlementaire. n° 476, nous proposons d'ajuster les dates des différentes périodes des CEE par coordination avec le principe d'une fixation par la loi, sur une base quinquennale, à compter de 2024, ainsi qu'avec l'annonce faite par le Gouvernement de prolonger d'un an la quatrième période. En conséquence, les prochaines périodes des CEE et leur mode de fixation seront les suivants : la période 2018-2020 est prolongée d'un an, jusqu'au 31 décembre 2021 et le volume d'obligations à réaliser demeure fixé par décret la période transitoire suivante, entre le 1 janvier 2022 et le 31 décembre 2023, verra son volume d'obligations être fixé par une loi ordinaire, avant la discussion de la première loi quinquennale toutes les périodes ultérieures, dont la première, entre le 1 janvier 2024 et le 31 décembre 2028, seront calées sur les périodes de la PPE et verront leur volume d'obligations déterminé par la loi quinquennale créée par le présent article.

Enfin, les certificats d'économies d'énergie ne seraient plus définis par la loi, alors que nous y sommes très attachés. Pour ces raisons, il n'est pas possible de conserver ces modifications.

mais pas de manière concomitante à son examen par le Parlement. Quant à l'amendement n° 204 rectifié, il tend à fixer des objectifs de CEE sur une période dix ans, contre trois ans actuellement, ce qui n'est pas souhaitable. En effet, une telle modification rendrait

partageons évidemment l'exigence de visibilité pour les acteurs, mais il ne nous semble pas souhaitable de fixer tous les objectifs des différents dispositifs dans la loi.

les preuves d'effets néfastes sur la santé liés à l'exposition aux émissions issues du trafic routier sont fortes. » Nous répétons à l'envi que des changements importants, pour ne pas dire radicaux, s'imposent dans notre société.

mais sûrement, vers le « tout voiture », encore et toujours. L'aspect de nos villes et de nos campagnes a-t-il changé à cet égard ? Non, nous sommes toujours dans le tout voiture, partout. Nous devons changer nos habitudes, et, j'ose le dire, revenir à des habitudes anciennes. Qui, très jeune, n'est pas allé à l'école à pied

donc prioriser la politique énergétique nationale pour répondre à l'urgence écologique et climatique. Les transports, responsables de plus du tiers des émissions de gaz à effet de serre en France, contribuent de manière importante aux changements climatiques. La transition vers des modes de transport plus sobres en énergie et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre doit être prioritaire. D'autre part, la lutte contre le réchauffement climatique passe également nécessairement

prévoit déjà de fixer des objectifs de développement des énergies renouvelables en matière de carburant, reprenant ainsi la terminologie de l'article L. 100-4 du code de l'énergie.

l'ensemble des objectifs que celle-ci doit fixer en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de réduction de la consommation d'énergie, de diversification de notre mix énergétique, notamment, participent tout à fait directement à l'adaptation de nos politiques publiques et de notre modèle économique au changement climatique. Je sollicite le retrait

d'atténuation et d'adaptation, comme c'est du reste mentionné dans le plan national d'adaptation au changement climatique. Cependant, les objectifs en matière d'énergie renouvelable ou d'émissions font l'objet de cibles chiffrées, ce qui justifie le principe d'une loi de programmation. L'adaptation,

De plus, sur la forme, la loi visée au présent article concerne les objectifs de politique énergétique et sera codifiée dans le code de l'énergie, ce qui n'est pas forcément l'idéal pour intégrer l'adaptation. Je vous propose donc de retirer cet amendement, qui me semble effectivement soulever des difficultés.

M. Bernard Buis. L'article 1 A prévoit que la loi fixera, pour deux périodes successives de cinq ans, les objectifs de développement, dans la consommation finale brute d'énergie, pour l'électricité, la chaleur, le carburant et le gaz. Toutefois, à la différence des autres énergies, les objectifs de développement des énergies renouvelables électriques sont actuellement définis en proportion de la production d'électricité. Afin de ne pas introduire de difficulté, il est proposé de supprimer les mots « dans la consommation finale brute d'énergie », pour que les objectifs puissent être définis comme aujourd'hui.

La France est sur la bonne trajectoire pour atteindre cet objectif, en majeure partie grâce à la contribution des biocarburants de première génération, qui repose sur les atouts de son agriculture et de ses territoires. La contribution fondamentale du secteur des transports à l'atteinte de l'objectif de neutralité carbone doit donc être affirmée par la loi de programmation énergétique.

amendement est satisfait par le texte adopté par la commission, qui prévoit que la loi quinquennale détermine des objectifs de développement des énergies renouvelables fixés par la loi quinquennale portant sur le carburant. Il vaut mieux utiliser le terme « carburant

puis, tous les cinq ans, afin de prendre en considération les enjeux liés au remplacement, au renouvellement et au recyclage des ouvrages, des infrastructures des équipements énergétiques. Il s'agit de mettre en oeuvre une politique écologique et climatique durable, compatible avec les exigences de préservation, de protection et de sauvegarde de l'environnement, des paysages et des sites. À cette fin, il faut anticiper le cycle de vie des ouvrages, infrastructures et équipements énergétiques.

premier ordre. Il est en lien avec le projet de loi. D'une part, les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d'énergie, modifiés par l'article 1, ne peuvent être atteints sans prendre en compte l'effet global des installations de production d'énergie, y compris celui qui est lié à leur démantèlement, sur ces émissions ou cette consommation. D'autre part, le recyclage est un objectif visé par la directive du 11 décembre 2018. En outre, des dispositions sur le recyclage figurent d'ores et déjà dans le projet de PPE, qui prévoit, pour les énergies renouvelables électriques, de « préparer le recyclage à grande échelle des installations en fin de vie

du Gouvernement ? La question du démantèlement et du recyclage des installations énergétiques est au coeur des préoccupations du Gouvernement. Toutefois, ces éléments sont d'ores et déjà intégrés dans les objectifs de développement des énergies renouvelables, puisque l'atteinte de ces derniers nécessite de renouveler une partie de nos installations de production. Je pense notamment au des éoliennes.

dans la loi fixant les priorités d'action et la marche à suivre pour répondre à l'urgence écologique et climatique, en 2023, puis, tous les cinq ans. commission ? Les objectifs figurant dans cet amendement seraient très éloignés de la politique énergétique puisqu'ils porteraient sur la préservation de l'environnement, des paysages et des sites. Le régime juridique applicable aux domaines précités relève d'ailleurs non du code de l'énergie, mais du code de l'environnement. Dès lors, il est préférable de ne pas intégrer à la loi quinquennale des dispositions qui feraient perdre de vue son objectif premier : la détermination des objectifs et des priorités d'action de la politique énergétique nationale.

fixés pour cinq ans, exprimés en millions de tonnes de CO2 équivalent. Actuellement, les émissions stagnent, voire repartent légèrement à la hausse. L'action doit donc être accélérée pour mettre le pays sur une bonne trajectoire. Nous proposons, par cet amendement, de fixer les budgets carbone

Aujourd'hui, les budgets carbone sont des outils sous-utilisés, car ils sont non contraignants. Il convient donc de faire passer le niveau de décision de la stratégie nationale bas-carbone dans laquelle est fixé le budget carbone, du décret à la loi, afin d'accroître sa valeur contraignante

sont aussi nombreux, c'est parce qu'en signant l'accord de Paris sur le changement climatique en 2015 presque tous les pays du monde se sont engagés à maintenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement au-dessous de 2 degrés par rapport au niveau préindustriel et à poursuivre l'action menée pour la limiter à 1,5. Pour y parvenir, la politique climatique française doit s'appuyer sur la stratégie nationale bas-carbone, la SNBC, qui définit les budgets carbone, soit les plafonds d'émissions de gaz à effet de serre à respecter dans tous les secteurs durant le quinquennat en cours et les deux suivants, selon une trajectoire dégressive. C'est ainsi que certains considèrent la SNBC comme plus importante que la PPE en raison de son effet structurant. Or, aujourd'hui, la programmation pluriannuelle de l'énergie, la stratégie nationale bas-carbone et les budgets carbone qui en résultent sont de nature réglementaire et échappent à la compétence du Parlement. Parlement. Élever la définition des budgets carbone au rang législatif leur permettrait d'avoir un effet plus contraignant et restaurerait pleinement le rôle du législateur par rapport au pouvoir réglementaire. Cet amendement répond aussi à une recommandation du Haut Conseil pour le climat, qui précise que « le niveau du budget carbone et sa répartition sectorielle devraient être fixés par la loi

Le cadre actuel est juridiquement et politiquement trop faible pour mener la France vers la neutralité carbone en 2050. » Elle ajoute à propos des budgets carbone tels que

La fixation des budgets carbone par la loi quinquennale n'est pas opportune. Tel qu'il a été adopté par la commission, l'article 1 A prévoit que la loi quinquennale détermine des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour trois périodes successives de cinq ans, les budgets carbone étant fixés par décret et devant être compatibles avec ces objectifs. Cela signifie que les amendements identiques sont déjà satisfaits ! Cette construction renforce substantiellement le rôle du Parlement dans ce domaine. Aller plus loin, en confiant au législateur le soin de déterminer les budgets carbone eux-mêmes, complexifierait l'édifice d'ensemble pour des bénéfices qui n'ont rien d'évident. En effet, nous entrerions alors dans des débats très techniques, exprimés en mégatonnes de CO2, alors que notre rôle me semble être de fixer une direction, un cap. Cela est d'autant moins souhaitable que le dispositif s'articulerait mal avec les autres outils de la compatibilité carbone. de même que le budget carbone sur le transport international ou l'empreinte carbone de la France- institués sous une forme indicative par les articles 1 B et 1 -sont

il est prévu que la loi de programmation quinquennale précise les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour trois périodes successives de cinq ans. Ensuite- ce paragraphe n'est peut-être pas très lisible -, le III du présent article fait le lien entre ces objectifs globaux et la prise en compte dans les budgets carbone de chacun des secteurs. De plus, l'adoption de ces amendements ferait perdre le fondement législatif de la déclinaison de ces budgets carbone au niveau de la SNBC.

Nous proposons de le faire maintenant, car le secteur du bâtiment doit déjà intégrer la réglementation thermique 2020. De surcroît, notre pays est prêt et nous avons vraisemblablement besoin d'indicateurs réactualisés et plus fiables pour affronter la résilience des populations.

pour figurer parmi les objectifs devant être fixés par la loi quinquennale. Au demeurant, l'objectif visé par les auteurs de cet amendement est pour partie satisfait par d'autres dispositions du texte. Ainsi, l'article 1 prévoit l'institution d'une « feuille de route

du Gouvernement ? Le Gouvernement partage l'importance accordée au confort d'été dans le contexte du changement climatique en cours, notamment pour la future réglementation sur les bâtiments neufs.

en pratiquant un dumping considérable sur les coûts de livraison des biens qu'elles commercialisent. C'est en partie ce qui explique qu'Amazon dégage un résultat net aussi faible en proportion de son chiffre d'affaires. la législation avait interdit la livraison gratuite, les plateformes ont réussi à la contourner en proposant une livraison à quelques centimes. Au-delà des contraintes de concurrence déloyale pour les commerces physiques,

et de consommation d'énergie des véhicules. Le présent amendement vise donc à interdire que le tarif de livraison d'un bien commercialisé par une entreprise de e-commerce soit inférieur à son coût économique.

il contraindrait les entreprises de commerce en ligne à intégrer dans leurs tarifs de livraison le coût social et environnemental induit par la consommation énergétique et les gaz à effet de serre émis par ladite livraison.

Si cet amendement semble aller dans cette direction, il présente deux écueils majeurs. Tout d'abord, le fait que cette obligation soit limitée aux commandes réalisées le e-commerce me semble poser un vrai un vrai problème de nature constitutionnelle. Par ailleurs, cette obligation soulève la difficulté de l'individualisation des coûts de livraison dans le cadre d'envois de produits massifiés. Finalement, la mise en place d'un dispositif tendant à responsabiliser les chargeurs et les consommateurs quant au coût du transport devrait, à mon sens, faire l'objet d'une réflexion d'ensemble sur les modalités les plus adaptées d'une meilleure fiscalité environnementale,

et je me tourne vers le rapporteur : nous sommes la chambre des territoires. Nous défendons les centres-villes et les centres-bourgs. Nous avons examiné une proposition de loi sur le développement du e-commerce et des grandes centrales

nationale, impose que la programmation pluriannuelle de l'énergie fasse l'objet d'une synthèse pédagogique accessible au public. Nous sommes favorables à cette disposition, qui permettra aux Français de mieux saisir les enjeux de notre politique énergétique, notamment en matière de lutte contre le changement climatique.

Vous n'avez pas oublié, mes chers collègues, que notre jeunesse a manifesté ces derniers temps, tous les vendredis, pour le climat et contre le désastre annoncé. Or nous voulons des citoyens éclairés et capables de faire des choix. La politique énergétique et la programmation pluriannuelle de l'énergie, sur laquelle elle se fonde, traitent, en effet, de sujets complexes, qui méritent d'être vulgarisés auprès du jeune public, afin, notamment, que ce dernier puisse être sensibilisé très tôt

D'autre part, le ministère de l'éducation nationale intègre déjà la lutte contre les changements climatiques et la promotion du développement durable dans le cadre des programmes scolaires. Huit axes de développement ont d'ailleurs été présentés par le ministre

Connaître les possibilités du territoire en matière d'ENR est, en effet, absolument fondamental pour prévoir le développement de celles-ci. Nous souhaitons cependant soulever quelques interrogations,

ces puits de carbone doivent être non seulement en nombre suffisant, mais également en bon état. Ainsi, outre les arbres, le volume de bois mort en forêt est nécessaire pour la biodiversité, elle-même nécessaire à leur conservation.

d'autres, nous plaidons pour une maîtrise publique qui nous semble absolument nécessaire. Nous ne sommes évidemment pas opposés au développement des ENR, bien au contraire, mais le climat et l'énergie ne peuvent être envisagés indépendamment de tout contexte et, notamment, des nécessités propres à la biodiversité.

Il est important que la programmation pluriannuelle de l'énergie précise les gisements disponibles pour les énergies renouvelables, afin de clarifier la définition des objectifs et des mesures à mettre en oeuvre, et que cette caractérisation soit soit la plus précise possible. Cependant, le concept de « zone géographique » est flou et n'apporte pas de précision utile à l'élaboration de la PPE. Il pourrait, en revanche,

Face à l'intermittence des énergies renouvelables et à leurs coûts de système, soulignés par l'OCDE, la France ne saurait sacrifier son énergie nucléaire pilotable, propre et compétitive, au profit du maintien des énergies fossiles carbonées. Alors que le nucléaire est une source d'énergie bas-carbone utile pour tendre vers un mix énergétique décarboné, il n'est pas concevable de réduire nos capacités de production nucléaire avant que ne soient mises à l'arrêt toutes nos centrales à charbon, lourdement émettrices de gaz à effet de serre.

Cela va mieux en le précisant Il a le mérite de rappeler que la transition énergétique ne peut se réaliser sans le recours à l'énergie nucléaire, qui constitue une source d'énergie largement décarbonée. Pour autant, l'élaboration d'une stratégie de démantèlement des installations relève de la responsabilité de l'exploitant, sous le contrôle de son autorité de régulation. Par ailleurs, le dispositif serait peu applicable, puisque la fermeture des quatorze réacteurs envisagée d'ici à 2035 ne doit pas conduire à la fermeture complète de centrales. Enfin, il est pour partie satisfait, puisque la commission a adopté le principe d'un ordre de sortie des énergies fossiles en précisant qu'« il est mis fin en priorité à l'usage des énergies fossiles les plus émettrices de gaz à effet de serre », au premier rang desquelles figure le charbon.

mesure est superfétatoire, puisque l'exploitant est déjà soumis à des obligations assez exigeantes : il doit présenter un plan pour atteindre atteindre les objectifs fixés par la PPE dans un délai maximal de six mois après l'approbation de celle-ci. L'article 1 du présent projet de loi prévoit d'ailleurs de renforcer ce dispositif, notamment en donnant la possibilité à l'autorité administrative de prononcer une mise en demeure, voire des sanctions, en cas d'incompatibilité. Dans le même ordre d'idées, l'initiative de la commission, l'article 1 a été complété par une « feuille de route relative aux opérations de démantèlement des installations nucléaires » annexée à la PPE qui contribuera, elle aussi, à mieux piloter les engagements pris. En outre, le plafond ainsi fixé est excessivement rigide, alors que le projet de PPE intègre plusieurs scénarios en termes de part de l'énergie nucléaire dans le mix électrique en 2028 et que le plafond actuel, plus élevé,

amendement vise à mieux anticiper ces fermetures en identifiant et en quantifiant les emplois directs et indirects

Comme le souligne très justement le rapport, nous ne disposons d'aucun élément substantiel sur les effets économiques et sociaux induits par l'arrêt envisagé de quatorze réacteurs d'ici à 2035.

C'est pourquoi, à nos yeux, il est impératif que le Parlement soit informé, à travers le plan stratégique d'EDF, non seulement des dispositifs mis en place pour les salariés affectés par les fermetures, mais aussi du volume d'emplois possibles supprimés au sein de l'entreprise, des effets sur les salariés des sous-traitants, des dispositifs d'évolution, de formation, ainsi que de l'utilisation et de la valorisation des compétences dans les nouvelles filières.

sur le dos des salariés d'EDF, des sous-traitants et de leurs compétences.

Vouloir aller au-delà et exiger qu'EDF soit comptable des suppressions d'emplois directs comme indirects serait déraisonnable et renverrait la balle à l'exploitant, alors que cette évaluation ressortit clairement aux services de l'État, qui est à l'origine de ces décisions. L'avis de

sur l'accompagnement des fermetures des centrales à charbon. Comme l'a indiqué M. le rapporteur, à l'exception de la centrale de Fessenheim, qui fait l'objet d'un contrat de territoire intégrant un ensemble de mesures spécifiques, les fermetures des prochains réacteurs nucléaires ne sont pas prévues dans un délai

la reformulation qui vise à intégrer les sous-traitants pourrait apparaître comme une avancée, mais sa rédaction pose beaucoup de questions. C'est pourquoi le Gouvernement y est également défavorable.

actions, en particulier, dans les domaines de la prévention et de la lutte contre la pollution de l'air, de la prévention de la production de déchets, du réaménagement et de la surveillance de certaines installations de stockage de déchets ultimes, de la réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et du développement des énergies renouvelables, notamment d'origine végétale. Sans oublier le développement des technologies propres et économes et la lutte contre les nuisances sonores. Vouloir élargir les missions de cet établissement à la lutte contre le réchauffement climatique nous paraît une pure déclaration d'intention,

d'empreinte carbone, en y intégrant, bien évidemment, les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation de biens et services sur le territoire national, mais aussi les exportations, voire les importations, afin de disposer d'une

ce dispositif conférerait à cet indicateur une portée prescriptive susceptible d'entraîner des effets juridiques non anticipés sur les documents de programmation et le soutien aux projets publics.

a déjà en partie eu lieu hier, je me permets d'insister sur l'importance du concept d'empreinte carbone et la nécessité pour la France d'être proactive dans la définition de celui-ci.

Ainsi, le corridor rhodanien, les accès aux grands cols alpins et pyrénéens, la traversée de l'agglomération lyonnaise et le périphérique parisien sont autant de goulets d'étranglement où s'observe une pollution quasi permanente due au flot incessant de poids lourds. Pourtant, des solutions alternatives existent. Inspirons-nous de nos voisins

ce ne peut pas être dans le cadre des modalités de calcul de l'empreinte carbone de la France. En effet, la finalité de cet outil est de nature objective, non prescriptive : il s'agit d'offrir une connaissance globale des émissions de gaz à effet

Cette loi devra préciser les modalités nécessaires à l'application de l'empreinte carbone de la France. la commission ? La loi quinquennale n'a pas à fixer de dispositions relatives à l'empreinte carbone, puisque le présent article prévoit qu'elles seront déterminées par décret. Par ailleurs, je répète que, faute d'être suffisamment encadré, cet indicateur reposant sur une méthodologie encore inaboutie pourrait avoir des effets juridiques non anticipés sur le contenu des documents d'urbanisme et le soutien aux projets publics. L'avis de

Il n'y a pas lieu, selon moi, de reporter à 2022 la prise en compte de l'empreinte carbone, sous le prétexte de difficultés méthodologiques. Dans son rapport sur les nouveaux indicateurs de richesse, publié en février 2018, l'Insee précise que l'empreinte carbone permet d'apprécier les pressions globales sur le climat de la demande intérieure française, quelle que soit l'origine géographique des produits consommés. L'empreinte carbone est donc un indicateur reconnu par les institutions françaises. Il est essentiel que, dès la prochaine stratégie nationale bas-carbone, des objectifs précis de réduction de l'empreinte carbone soient fixés.

elle s'appuie sur de nombreuses estimations, et les données définitives ne sont arrêtées que quatre ans après l'année concernée. Pour définir des objectifs robustes et crédibles, il faut travailler plus en profondeur sur la méthode et sur l'évolution quantitative de l'empreinte carbone dans les prochaines années.

Cet article nous paraît particulièrement intéressant, dans la mesure où il prévoit que le Gouvernement devra remettre au Parlement, chaque année à partir du 1 octobre 2019, un rapport sur la compatibilité du projet de loi de finances avec l'objectif international de limitation du réchauffement climatique, en considérant les impacts positifs et négatifs.

Cela semble logique, puisque cette évaluation sera établie au regard des engagements pris par la France en matière d'émissions de gaz à effet de serre aux plans national et international. Je le dis sans esprit de polémique : heureusement qu'un tel rapport n'a pas été annexé à la dernière loi de finances, qui nous a placés encore très loin des objectifs de transition écologique

Je pense également aux engagements de ratification de traités particulièrement incompatibles avec nos engagements climatiques liés à la COP21 et à l'accord de Paris- nous en avons largement débattu. Je pense enfin à votre politique en matière de transport ferroviaire, qui conduit à mettre chaque jour un peu plus de camions sur les routes : casse du fret ferroviaire, abandon des petites lignes autres désengagements des pouvoirs publics. Et que dire de la suppression de plus de 800 postes en 2018 au sein du ministère de l'écologie ? Du gel des crédits à hauteur de 115 millions d'euros ? Ce rapport devra aider à passer des paroles aux actes, faute de quoi son utilité sera grandement limitée. Pour aller plus loin, nous considérons que non seulement la loi de finances, mais l'ensemble des projets de loi devraient être abordés sous le prisme des problématiques liées à la transition écologique. Le Haut Conseil pour le climat demande d'ailleurs que l'ensemble des projets de loi soient examinés en fonction de leur compatibilité avec la stratégie nationale bas-carbone et les quotas qui y sont définis.

durable ? La France s'est engagée, comme les autres pays du monde, à atteindre les objectifs de développement durable, ou ODD, fixés par les Nations unies pour 2030. Il paraît essentiel de mieux intégrer la prise en compte de ces objectifs dans l'élaboration et le vote du budget, qui détermine les politiques publiques mises en oeuvre et financées dans l'année à venir, comme l'ont fait d'autres pays européens.

solaire. La réflectance d'une paroi ou d'une toiture est idéale pour isoler des fortes chaleurs. Il faut pouvoir utiliser des dispositifs variés pour améliorer l'efficience thermique de nos bâtiments.

Nous sommes donc consultés plus de sept mois après la décision ... Faut-il rappeler que le Parlement n'est pas une simple chambre d'enregistrement de la volonté présidentielle ? Très bien ! Alors qu'existent déjà le Commissariat général au développement durable, durable, le Conseil national de la transition écologique et le Conseil de défense écologique et que l'Ademe intègre à présent la lutte contre le réchauffement climatique, nous pouvons nous interroger sur la pertinence de la création d'une nouvelle instance.

Certes, le Haut Conseil pour le climat est composé d'experts plutôt que de ministres, et il s'agit d'un organe dit indépendant dont le premier rapport s'est révélé extrêmement critique. Reste que la multiplication d'instances consultatives, donc de rapports et d'avis non contraignants, n'engage pas les politiques publiques menées par le Gouvernement ni ne constitue une mise en actes des discours tenus sur l'urgence climatique. La prise en compte des avis du Haut Conseil pour le climat par les collectivités territoriales est proposée à l'article 2 , et le Gouvernement devra présenter retours et justifications sur les rapports. Toutefois, cela ne signifie en rien qu'il suivra effectivement et activement les recommandations émises. Enfin, ces instances isolées, centrées sur le climat et le réchauffement climatique, entretiennent la sectorisation des problématiques environnementales, comme s'il s'agissait de politiques publiques pouvant être menées indépendamment les unes des autres. L'urgence en impose au contraire une prise en compte totale et transversale. Ainsi,

qui consiste à faire du Parlement une chambre d'enregistrement et à placer la représentation nationale devant le fait accompli. Désormais, le Gouvernement prend des décrets avant de faire ratifier ceux-ci par la loi. C'est le monde à l'envers

le Haut Conseil pour le climat, le Conseil national de l'air, le Conseil national de la transition écologique, le Conseil supérieur de l'énergie. Peut-être faudra-t-il un jour rationaliser ces instances,

tendant à concilier la vision politique et l'expertise scientifique, je m'interroge, madame la ministre : en quoi la multiplication de ces instances facilite-t-elle la prise en compte des sujets traités ? Est-ce une démarche de simplification ? On parle beaucoup d'agilité, de fluidité. Le Haut Conseil pour le climat y participe-t-il ? Enfin, comment cette instance va-t-elle articuler son action dans le processus démocratique, entre les temps du diagnostic, de l'expertise, le travail du

dernier par une décision du Président de la République ? Au-delà de la forme contestable, sur le fond, nous sommes favorables à l'existence du Haut Conseil pour le climat, qui a d'ores et déjà rendu un avis très intéressant.

Nous vous proposerons un amendement en ce sens. Plus fondamentalement, et c'est l'objet de sa recommandation n° 4, le Haut Conseil estime que la transition bas-carbone doit être juste et perçue comme telle, pour que les actions soient durablement soutenues par l'ensemble de la société.

Voilà qui sonne comme une remise en cause des politiques gouvernementales, qui n'ont fait que renforcer jusqu'à présent les inégalités sociales, ce qui a d'ailleurs conduit au mouvement des gilets jaunes. La parole est à M. Ronan Dantec, sur l'article.

Or, vous le savez, les émissions de gaz à effet de serre sont reparties à la hausse l'année dernière. La situation est très préoccupante. Le rapport que le Haut Conseil vient de rendre prouve son indépendance. Espérons qu'il sera entendu, espérons que vous l'entendrez, madame

Aujourd'hui, il n'est, en effet, plus possible de dissocier les défis majeurs liés aux gaz à effet de serre de ceux des polluants de l'air. Les scientifiques se doivent de travailler conjointement sur ces deux sujets dont les enjeux sont intimement liés. L'amendement n° 178, présenté

à commencer par l'effondrement du vivant et la sixième extinction des espèces du fait des activités humaines. Les interactions et rétroactions entre bouleversement du climat et destruction de la biodiversité sont telles qu'une approche intégrale et systémique des enjeux écologiques est absolument impérative dans l'expertise apportée

est à Mme la ministre. Le présent amendement vise à supprimer la soumission du projet de programmation pluriannuelle de l'énergie à l'avis du Haut Conseil pour le climat. En effet, les dispositions qui relèvent de la compétence du du Haut Conseil sur les volets de la politique énergétique sont déjà intégrées dans la SNBC, sur laquelle cette instance rend obligatoirement un avis. Les remarques qui devront être intégrées à la SNBC seront donc nécessairement prises en compte dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, puisque celle-ci doit être compatible avec la SNBC. De plus, le Haut Conseil peut également se saisir sur sa propre initiative des questions relatives à son domaine d'expertise. Par conséquent, il peut s'il le souhaite émettre un avis sur la PPE. madame la rapporteure Or le Haut Conseil pour le climat a vocation à rendre des avis sur les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il ne semble pas opportun d'élargir son champ de compétences à la qualité de l'air.

et décline de manière plus opérationnelle que cette dernière l'avenir de notre politique énergétique filière par filière. Il me semble donc impératif d'avoir un avis du Haut Conseil sur cette programmation. C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable

d'experts en matière de changement climatique. Il est d'ores et déjà prévu que le Haut Conseil dans ses rapports annuels analyse plus largement l'incidence environnementale des politiques publiques en faveur du climat. C'est dans ce cadre qu'il pourra mettre en évidence les synergies et, le cas échéant, alerter sur des incohérences entre politiques publiques. Un élargissement du champ à une problématique spécifique, mais plus large, risquerait de nuire à l'objectif principal de

sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, sur le développement des puits de carbone et sur la réduction de l'empreinte carbone. À ce titre, il rend des rapports. Il comprend au plus douze membres choisis en raison de leur expertise scientifique, technique, économique dans le domaine des sciences du climat.

la lecture de. Les écosystèmes et la nature en général sont des alliés à ne pas négliger dans notre lutte contre le changement climatique. Les écosystèmes les plus vulnérables ont d'ailleurs été répertoriés : ce sont les zones arctiques montagneuses, la forêt amazonienne

Il est par exemple important que cette instance compte parmi ses membres des experts en matière d'agriculture, de sols, de forêts compte tenu du rôle majeur joué par ces derniers sur les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre.

Antiste. Les territoires ultramarins, majoritairement insulaires et situés en zone tropicale, sont particulièrement confrontés aux conséquences du réchauffement climatique et à la montée des eaux. Les événements récents aux Antilles ont mis en exergue la fragilité et l'exposition de ces territoires.

un des experts nommés au Haut Conseil pour le climat le soit en raison de son expertise dans les problématiques liées aux incidences du réchauffement climatique dans ces territoires.

Antiste. Si la modélisation du climat dans les zones d'outre-mer reste encore un domaine de recherche très jeune, les grandes tendances de l'évolution du climat sont mieux connues aujourd'hui, à l'exception de ce qui se passe dans les très petites îles. Il est donc nécessaire d'évaluer précisément et particulièrement pour ces régions souvent îliennes, où l'interconnexion énergétique n'est pas possible,

durable ? Cet amendement vise à inclure dans le rapport annuel du Haut Conseil un volet relatif au développement et à la sécurité d'approvisionnement énergétique par les énergies renouvelables en outre-mer en corrélation avec les évolutions climatiques. Or la vocation première du Haut Conseil est d'émettre un avis sur les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'une manière générale. Il ne semble donc pas opportun d'ajouter un tel volet dans le rapport annuel, d'autant que celui-ci est éloigné des missions du Haut Conseil. La commission émet un avis défavorable

Antiste. Pour les raisons susvisées, il paraît légitime que le rapport du Haut Conseil pour le climat s'intéresse à l'impact des politiques publiques sur les territoires ultramarins.

Il nous faut augmenter le nombre des pistes cyclables, qui ne sont pas toujours bien accueillies et qui sont pourtant nécessaires. Il nous faut revoir l'organisation de nos villes, de nos centres-bourgs, réinventer les usages. Un état des lieux doit être réalisé pour lever ces freins. Les rapports du Haut Conseil doivent impérativement se pencher sur la mobilité douce, car c'est un levier puissant de progrès dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

toutes les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il n'est donc pas nécessaire de préciser qu'il devra notamment porter sur le développement des mobilités décarbonées. Si l'on voulait entrer dans ce niveau de détail, il faudrait être beaucoup plus exhaustif

Nous considérons que l'on ne peut plus aujourd'hui dissocier les enjeux climatiques et écologiques des grands choix économiques et budgétaires. La préservation du climat et du vivant doit au contraire être au centre des orientations des politiques économiques et s'appuyer sur une trajectoire financière. Nous avions d'ailleurs proposé que le Gouvernement lève un emprunt pour financer la transition énergétique. Nous sommes de ceux qui pensent que les grands investissements favorisant la transition écologique ne devraient pas être comptabilisés dans les critères de Maastricht. Il convient que le rapport annuel du Haut Conseil pour le climat soit transmis à la commission du développement durable,

celle-ci est limitée au Gouvernement, au président de l'Assemblée nationale, à celui du Sénat, et au président du Comité économique, social et environnemental. Autant dire qu'il s'agit d'un nombre extrêmement limité de personnalités, dont au moins deux sont très directement liées aux politiques mises en oeuvre par la majorité.

durable ? L'article 2 prévoit d'ores et déjà que le Haut Conseil puisse être saisi par le Gouvernement, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le président du CESE, ou encore s'autosaisir.

À mon avis, ce qui est beaucoup plus important, c'est que l'on inscrive bien dans la loi l'indépendance du Haut Conseil pour le climat. En effet, il n'est pas question ici de minimiser l'importance du réchauffement climatique et de réduire l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

En effet, il est essentiel que le Gouvernement introduise dans ce texte les éléments du tout premier avis du Haut Conseil, faute de quoi la crédibilité de celui-ci sera durement entamée et il sera réduit à un « machin » supplémentaire. En confiant cette mission au Haut Conseil pour le climat, sous réserve qu'il dispose des moyens adéquats, il s'agit également d'organiser une étude indépendante du Gouvernement sur la conformité des politiques menées par celui-ci avec ses engagements climatiques, notamment la stratégie nationale bas-carbone. Une telle expertise nous semble indispensable.

en conditionnant la soumission d'un projet ou d'une proposition de loi au respect de l'avis du Haut Conseil pour le climat, qui n'est qu'un organe consultatif. Le sous-amendement n° 487 du Gouvernement, quant à lui, vise à supprimer cette contrainte pour conserver uniquement la mention selon laquelle le Haut Conseil

à contribuer en fonction de leur potentiel à l'effort national. Le Haut Conseil pour le climat pourra apporter sa contribution à ces échanges. Il devra en particulier évaluer l'adéquation entre les politiques décidées et mises en oeuvre par les collectivités et les objectifs climatiques.

Or, dans le Sraddet, les éléments opposables sont toujours issus d'une norme ou d'une décision comportant des effets juridiques. En revanche, il existe un vecteur pertinent pour assurer le lien entre les avis du Haut Conseil pour le climat et l'élaboration du Sraddet : c'est le dispositif du « porter à connaissance